La séance est reprise. Mes chers collègues, je vais commencer par les « bonnes » nouvelles- j'insiste sur les guillemets ... Par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande l'inscription, le vendredi 8 mai au soir et le samedi 9 mai au matin, sous réserve de leur dépôt, des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Par ailleurs, en cas de nouvelle lecture de ce texte, il en demande l'inscription le dimanche 10 mai après-midi.

En cas de nouvelle lecture, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance serait fixé à l'ouverture de la discussion générale, comme il est de tradition.

Si même en France la censure sur les réseaux sociaux est monnaie courante, il semble que la fascination pour les solutions de facilité autoritaires et liberticides soit l'apanage de cet état d'urgence. Aujourd'hui, on nous propose de mettre en place un système d'information et de ciblage la localisation de nos téléphones, en ponctionnant nos données personnelles auprès des opérateurs. À une époque pas si lointaine, on aurait été scandalisé d'une telle menace potentielle pour nos libertés publiques. Mais, comme le dit Saint Augustin, à force de tout voir, on finit par tout supporter ... À force de tout supporter, on finit par tout tolérer ... À force de tout tolérer, on finit par tout accepter ... À force de tout accepter, on finit par tout approuver ! » Je serais tenté d'ajouter : Plutôt que de traquer nos compatriotes, le Gouvernement devrait se contenter d'assurer la sécurité informatique des citoyens, entreprises et institutions qui ont basculé vers le télétravail pour pouvoir se confiner. L'état d'urgence doit être également profitable pour garantir la cybersécurité dans le pays et renforcer notre prévention dans ce domaine. Comme le préconise la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), adoptons une stratégie globale, au lieu d'abandonner chacun à lui-même. Pour défendre les libertés publiques tout en combattant la propagation du virus, la priorité sur laquelle tout le monde est d'accord- ou devrait l'être -est de fournir aux Français les masques et tests de dépistage qui leur permettront de reprendre une vie normale

de rejeter ces amendements, pour une raison très simple : il nous paraît indispensable de donner à l'État la capacité

sur la base de l'identification de nos concitoyens qui auront été en contact avec des porteurs du virus. La tâche est titanesque.

le plus tôt possible : car chaque jour de perdu, ce sont des contaminations supplémentaires. Le caractère massif massif de ce système d'information centralisé doit répondre au caractère massif de l'épidémie. Il n'y a pas de déconfinement possible si la France n'est pas en mesure de procéder à cette identification des personnes ayant été en contact avec des porteurs du virus. Le texte dont nous débattons n'est porté à notre connaissance de législateur que pour une seule et unique raison : avec tant de personnes à contacter,

droit. Le Gouvernement pourrait fort bien mettre en place un système d'information centralisé sans le législateur. Le règlement général de protection des données (RGPD) que nous avons transposé dans la loi française l'y autorise, car son article 9 prévoit des dérogations au principe selon lequel on ne doit pas procéder à des traitements nominatifs de données de santé, des dérogations claires et destinées à servir un intérêt majeur majeur de santé publique. Or si nous ne sommes pas en présence d'un intérêt majeur de santé publique, je n'ai rien compris à la situation dans laquelle se trouve actuellement notre pays ... La question du recours

de l'obligation de secret à d'autres personnes que les médecins. Car il va de soi que les agents de l'assurance maladie qui concourront au bon fonctionnement du dispositif seront eux aussi assujettis au secret- mais pas le secret du médecin. sont les raisons pour lesquelles je demande au Sénat de ne pas adopter ces amendements.

L'autre système, de nouvelle génération, sera StopCovid. Cher Philippe Bonnecarrère,

L'intention du législateur sera déterminante pour que le Conseil puisse en apprécier exactement l'utilité et le mode opératoire.

d'ailleurs fait dans un contexte international particulier : il était utile de montrer qu'un continent entier se dotait d'un cadre juridique extrêmement protecteur des données personnelles, de la vie privée et des libertés publiques au moment même où les États-Unis,

Son décret d'application permet aux pouvoirs publics de mettre en place d'urgence des mesures de prévention individuelle et collective et, le cas échéant, de déclencher des investigations pour identifier l'origine de la contamination ou de l'exposition. Ce régime organise des mesures d'investigation et d'intervention et la collecte de toutes les informations indispensables pour la mise en oeuvre des mesures de prévention individuelle et collective. On voit que son champ d'application est extrêmement large et qu'il donne énormément de pouvoirs à l'État. Tout ce processus est bien évidemment fondé sur un traitement informatisé des informations de santé, qui a été validé par la CNIL à plusieurs reprises.

Nous avons donc là un dispositif parfaitement connu, éprouvé, encadré, respectueux des libertés individuelles, sur lequel la CNIL a déjà eu l'occasion de donner son avis. Je vous pose de nouveau la question, monsieur le ministre

a un fondement juridique qui se révèle à l'examen inapproprié pour ce que nous avons besoin de faire : remonter la filière des contaminations pour le Covid-19. C'est un système assez artisanal. Normalement, les informations sont anonymes. En fait, elles ne le sont pas,

des maladies à déclaration obligatoire, qui a besoin d'un certain toilettage si nous voulons qu'il fonctionne correctement. Monsieur Bonnecarrère, je suis d'accord avec vous

intéressant. Je pense que nous avons effectivement tout intérêt à développer la recherche épidémiologique sur la base de données anonymisées pour le Covid-19.

épidémiologique permettant de mieux connaître le virus, à travers l'examen de la situation médicale d'échantillons suffisamment nombreux de porteurs du virus et de patients. En tout état de cause, cher Philippe Bonnecarrère,

évoqué la possibilité d'intégrer le Covid-19 dans la liste des maladies à déclaration obligatoire. Nous n'avons pas retenu cette option, parce que nous pensons

et l'impérieuse nécessité de respecter la vie privée et les libertés publiques. Chacun a au fond de lui ces différentes exigences.

est notre position. Elle n'est pas majoritaire, mais nous avons tenu à en faire part au Sénat. Un certain nombre de nos collègues ont fait valoir la position de la commission des lois et de la commission des affaires sociales dans leur majorité

Je reconnais qu'il est peut-être inhabituel de présenter les choses ainsi, mais l'engagement politique n'a de sens que si l'on respecte le parler vrai. L'amendement

Cet amendement tend à encadrer les finalités auxquelles sont destinées la création d'un système d'information et l'adaptation des systèmes d'information existants, conformément à l'intitulé du chapitre II

non astreignant de la CNIL comme garde-fou, le Gouvernement démontre sa volonté de légiférer en solitaire sans accepter que sa prise de décision soit pondérée par les experts. À cet égard, j'avoue qu'il y a eu quelques évolutions depuis deux jours. La création d'un fichier recensant nos concitoyens n'a rien d'anodin ; l'histoire nous l'a bien démontré. Si un tel dispositif devait voir le jour, il semble impératif que de nouvelles précautions soient prises pour encadrer les atteintes disproportionnées aux données personnelles de nos concitoyens. Nous proposons donc par cet amendement de faire en sorte que tout prélèvement de données ne soit réalisé qu'avec le consentement de la personne porteuse du virus. Il paraît évident qu'il faille consulter le citoyen avant que ces informations privées ne soient transférées aux autorités alors même qu'elles devraient relever du secret médical. Bien que nous soyons opposés par principe à un système de prélèvement des données dans un objectif de fichage, semble qu'un droit de regard préalable du malade concerné permettrait de tempérer un dispositif qui serait uniquement régulé par les autorités ; cela créerait une relation de confiance. L'amendement Cet amendement, qui est présenté par l'ensemble de mon groupe, vise à obtenir le consentement des intéressés pour figurer dans ce que l'on nous a présenté tantôt comme un fichier, tantôt comme un système d'information ; tout le monde a bien compris que c'était la même idée. nous sommes favorables aux équipes épidémiologiques de terrain pour faire le travail tendant à casser les chaînes de contamination, autant nous considérons

Dans un souci d'efficacité, vous ne pouvez pas nous demander en plus de faire survivre ce système à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

refusent de prêter leur concours à ce qui est de nécessité publique : remonter les filières de contamination pour protéger nos concitoyens. C'est la raison pour laquelle l'avis des deux commissions- je me permets de le dire au nom de mon excellent collègue Alain Milon, mais il pourra le faire lui-même -est défavorable sur ces

J'évoque ce point, car Philippe Bas, avec cette ironie mordante qui nous fait souvent sourire, n'avait peut-être pas pris suffisamment au sérieux

prononcés mardi dernier à l'Assemblée nationale : « Notre politique repose, à cet égard, sur la responsabilité individuelle et sur la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l'égard des autres. »

spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant. La prise en compte du consentement serait de nature, selon moi, non pas à complexifier les procédures, mais au contraire à expliquer la démarche et la finalité

point de vue, il fut désagréable de lire, hier, que le chef de votre parti avait trouvé utile de qualifier le Sénat d'« irresponsable ». En effet, nous aurions eu le mauvais goût de ne pas cacher aux Français que nous ne sommes pas toujours d'accord avec votre méthode,

par exemple parce qu'il est malade, refuse de prêter son concours à la recherche des personnes qu'il a rencontrées et pu contaminer, c'est très grave

entre autres, d'un certain nombre de principes fondateurs du droit de la santé, en particulier le secret médical, lequel- je le rappelle -est non pas simplement une obligation déontologique pour les médecins, mais aussi, et avant tout, un droit des patients. Il est nécessaire Il est nécessaire de lever le secret médical pour instaurer ce système. Pour autant, il nous semble utile de prévoir un certain nombre de contrôles, de verrous, et de conserver l'esprit du droit de la santé,

vise à étendre la durée limite de conservation des données collectées dans le nouveau système d'information aux données partagées. L'amendement n° 48 n'est pas soutenu.

Monsieur le ministre, nous ne voulons pas vous donner un blanc-seing pour rédiger votre décret comme vous l'entendrez !

Certaines caractéristiques se dégagent cependant. Afin de permettre la détection des chaînes sociales de contamination, le projet de loi prévoit la création d'un système d'information qui comporterait des données de santé et d'identification. La collecte de ces informations devrait ensuite servir à déterminer les personnes ayant été en contact avec les malades, afin de tuer dans l'oeuf toute propagation du virus. Pour ce faire, ces données devront être accessibles à des agents agréés, notamment au sein des ministères. À de nombreux égards, cet article 6 est problématique ; tout le monde l'a plus ou moins reconnu. Il l'est, tout d'abord, car il permet la collecte de données privées. La CNIL nous a d'ores et déjà alertés sur les dangers que pourrait entraîner la création d'une liste des personnes malades. Rien ne permet en effet de garantir que des mesures coercitives et discriminatoires ne seront pas prises à l'encontre de ces dernières dans le but de contenir la pandémie. De plus, le fait que ces données médicales soient transmises à des membres du personnel des ministères porte atteinte au principe général et absolu du secret médical, qui est un élément fondateur et primordial de notre droit de la santé. Enfin, rien dans la rédaction du projet de loi ne garantit l'anonymisation des personnes malades susceptibles de pâtir d'une utilisation ultérieure du fichier constitué. Mes chers collègues, la santé publique est l'affaire de tous, elle est notre objectif commun, mais il ne saurait être atteint au prix de la diffusion de certaines de nos données certainement pas au détriment du secret médical. Le présent amendement vise donc à expurger l'article 6 de sa substance la plus attentatoire à la vie privée de nos concitoyens. L'amendement

Cet amendement vise à permettre la transmission à certains organismes de données nécessaires à l'accompagnement social des personnes vulnérables, dans le cadre des mesures prises pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Ces organismes peuvent en particulier être les services des collectivités territoriales,

Il est de fait important, dans le cadre du suivi des personnes qui ont été exposées à un risque de contamination, de savoir que leur premier test de dépistage a été négatif. Il faut cependant continuer de les suivre,

d'ailleurs d'encadrer le recours à des traitements algorithmiques pour certains actes de santé et pose une obligation d'information préalable du patient

amendement : « L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces systèmes d'information. « Chaque semestre à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé sur l'application des dispositions du présent article.

Je précise qu'on relève, dans l'exercice du pouvoir réglementaire, d'autres cas connus de lien entre l'avis conforme d'une autorité administrative indépendante

monsieur le ministre,

Cet amendement a été déposé très tard ; il n'a donc pas pu être examiné par la commission. Il vise à rappeler le caractère obligatoire de la transmission des informations collectées à chaque échelon de la chaîne de suivi des contacts. Nous avons du mal à interpréter cet amendement dans toute sa complexité. Peut-être M. le président de la commission des affaires sociales pourrait-il nous donner son sentiment à

bien au-delà de 100 000. Cela, c'est la théorie. Plus précisément, comme vous le savez, nous avons organisé le suivi épidémiologique en trois niveaux. Le premier niveau est assuré par les médecins de terrain, de premier recours : le médecin généraliste, le pneumologue,

apporter toutes les garanties nécessaires pour que cette infrastructure numérique, si elle est mise en oeuvre, puisse protéger les libertés individuelles. La parole

de risques supérieurs à ceux de départements similaires. C'était notamment le cas du Lot, du Cher et de la Haute-Corse, mais aussi de la Nièvre. S'agissant de ce dernier département, la surprise fut importante, car les chiffres du groupement hospitalier de territoire

celle d'une campagne aux espaces ouverts et à la densité faible qui protège sa population des conséquences, notamment sanitaires, auxquelles sont confrontées les populations vivant dans les zones de fortes concentrations humaines.

pour que l'élection des maires et des adjoints dans les communes ayant un conseil municipal complet ait lieu avant la fin du mois de mai.

Compte tenu de la situation spécifique des outre-mer, la lutte contre la propagation du virus passe de manière importante par les contrôles sanitaires aux frontières, en complément du confinement et de la montée en puissance des capacités sanitaires. C'est pourquoi une quatorzaine stricte est mise en oeuvre dans ces territoires en complément d'interdiction forte sur les mouvements de personnes vers ces territoires. Dès lors, et afin de s'assurer de l'effectivité de la quatorzaine préventive, il est proposé que ce soit le représentant de l'État qui détermine le lieu de réalisation de la quarantaine.

regrettant « la démarche irresponsable qui a conduit une majorité de sénateurs à ne pas voter en faveur de la déclaration du Premier ministre plaçant la logique politicienne avant l'intérêt supérieur du pays.

irresponsable dans notre démocratie, dans un État de droit, de considérer la contradiction démocratique comme un danger pour le bon fonctionnement de la Nation. Il s'agit d'une vision autoritaire d'un pouvoir qui un jour connaîtra l'opposition.

tant que lanceurs d'alerte sur la gestion globale de cette crise sanitaire et sur la stratégie de déconfinement. C'est notre droit, tout comme de déposer

sous la V République ! Nous avons donc pris nos responsabilités en vous accordant ce pouvoir qui pourrait être considéré dans d'autres Républiques comme exorbitant du droit commun. Mais nous avons mis un point d'arrêt ce soir

recours que nous porterons devant le Conseil constitutionnel, dans son immense majorité, le groupe socialiste et républicain s'abstiendra sur ce texte.

Je veux saluer, au nom de l'ensemble des sénatrices et sénateurs du groupe Les Républicains, les travaux de la commission des affaires sociales et de la commission des lois dirigés par leurs présidents, Alain Milon et Philippe Bas. ces deux jours, nous avons longuement débattu de la question de la responsabilité dans la mise en oeuvre du déconfinement. Artisans, petits commerçants, chefs d'entreprise, directeurs d'école, inspecteurs de l'éducation nationale, maires, en particulier ceux des petites communes, présidents de syndicat ou d'intercommunalité, tous ont et

pour assimiler les normes et les protocoles, urgence pour les mettre en oeuvre. Chacun est prêt à prendre un risque, afin de permettre une reprise progressive et sécurisée de l'activité économique,

Le Président de la République et le Gouvernement répètent quotidiennement qu'ils font confiance aux élus, aux maires en premier lieu, et à la société, mais faire confiance, c'est donner des garanties pour réassurer cette confiance. C'est pour cette raison que le Sénat a voulu clarifier le régime de responsabilité. Il souhaite cette clarification, parce que dans une situation exceptionnelle c'est d'abord au législateur de dire le droit, de fixer la règle et de lever les incertitudes juridiques liées aux interprétations à venir des juges. Il ne s'agit en aucun cas d'exonérer les maires, les directeurs d'école ou les chefs d'entreprise, puisqu'un régime de responsabilité demeure. Il s'agit encore moins d'exonérer le Gouvernement et la haute administration de leurs responsabilités. Il s'agit, contrairement aux déclarations d'une cabale qui ne prospèrera pas, de protéger les petites mains opérationnelles du déconfinement, celles qui vont mettre en oeuvre les protocoles qu'elles n'ont pas préparés, pour lesquels elles n'ont pas été consultées et qu'elles déclineront par sens du devoir.

et, dans un temps limité, d'encadrer et de préciser la responsabilité de chacun. C'est la clé de l'engagement dans la confiance. Le texte consensuel de la commission, gravé dans le marbre par le vote unanime contre l'amendement de suppression, est un message fort du Sénat, toutes tendances politiques confondues. Le deuxième apport essentiel de la commission concerne le dispositif de traçage. Nous l'avons dit sur ces travées, casser une chaîne de transmission au XXI siècle passe par un dispositif de traçage de notre temps, mais sécurisé. C'est la clé d'une stratégie plus offensive pour casser les reins de cette épidémie. L'outil numérique est le plus simple et le plus efficace pour vaincre.

Elles constituent des garde-fous essentiels. En conclusion, le groupe Les Républicains votera pour ce texte largement amendé en première lecture. Nous demeurerons attentifs à ce que les apports du Sénat ne soient pas dénaturés lors de la navette parlementaire qui pourrait être source d'améliorations bienvenues, mais qui ne saurait être l'occasion de balayer les apports de notre Notre bienveillance sera à la hauteur de la prise en compte de ce travail que nous avons voulu concret et précis et dont nous espérons que la navette parlementaire saura tirer le meilleur profit. Cela conditionnera la position future de mon groupe.

nous ne sommes pas en guerre et, en fait, c'est peut-être pire, pour reprendre les mots de Régis Debray : « En fait, une catastrophe, c'est pire. Dans une guerre, on meurt pour quelque chose et il y a deux camps. Mais un virus est neutre et tout le monde est contre. Le Covid-19 n'a ni drapeau, ni haine, ni but de guerre. Le tragique, le douloureux, c'est l'absence de sens, et donc l'absurde.

Ce qui nous était demandé au mois de mars et, plus encore, ce qui nous est demandé aujourd'hui est presque d'ordre anecdotique, tant le champ des décrets et des ordonnances ouvert au Gouvernement est large et tant les mesures réglementaires seront décisives dans la gestion de la crise. nous comprenons l'urgence à agir et les circonstances exceptionnelles dans lesquelles il nous est demandé de légiférer, mais comment ne pas s'interroger sur le peu de cas qui est fait du Parlement,

alors que dans les transports espagnols les policiers distribuent des masques gratuitement, avec ce projet de loi, vous nous proposez d'étendre les pouvoirs de police aux agents des transports publics et vous retoquez notre proposition visant à rendre gratuits les masques qui seront pourtant obligatoires dans les transports. D'autres mesures étaient possibles, mais les choix se sont portés sur une gestion de la crise sanitaire par des mesures de police administrative coercitive, les amendements déposés par le Gouvernement ayant confirmé nos craintes. Coercition à tout va, c'est donc une priorité du Gouvernement, alors que alors que la vérité est ailleurs, oserais-je dire. Cette réalité, c'est le manque de masques, l'insuffisance de tests, l'impréparation des transports publics, les difficultés de l'école à reprendre après des années de disette budgétaire ... La réalité, monsieur le ministre, c'est la crise sociale dramatique qui s'annonce, alors que déjà la faim gagne nombre de familles devant les soupes populaires. Nous avons fait un certain nombre de propositions, afin d'améliorer les conditions de vie largement dégradées de nos concitoyens : garantie du libre choix des parents pour ce qui concerne la reprise ou non de l'école par leurs enfants, interdiction des licenciements durant cette période de crise, interdiction des expulsions locatives,

! S'agissant des autres mesures contenues dans ce texte de prorogation, le dispositif de mise en quarantaine n'est pas encadré dans le respect des droits fondamentaux ; il n'y a par exemple aucune précision concernant le lieu de placement en quarantaine ou à l'isolement. Tout ne Tout ne peut pas être renvoyé au règlement, comme nous l'a indiqué le Défenseur des droits. Il en est de même pour l'article 6 qui a été adopté.

d'abord, la notion de recueil volontaire des données, pourtant essentielle et exigée par le règlement européen de protection des données ; ensuite, l'anonymisation qui n'est pas garantie- au contraire, le fichier est nominatif. Finalement, les garanties qui avaient été annoncées dans le cadre du projet StopCovid, projet bien contestable par d'autres aspects, sont donc absentes de ce projet final. Enfin, sur les questions de responsabilité, nous l'affirmons clairement, les maires ne doivent pas subir les conséquences des défaillances graves de l'État dans la gestion de la crise sanitaire. Pour autant, nous refusons tout élargissement incontrôlé de la déresponsabilisation. Nous l'avons expliqué, la lutte contre l'épidémie peut se poursuivre en dehors d'un état d'urgence ; cela permettrait de renforcer l'effort commun et la mobilisation générale. Le Parlement devrait voter son arrêt pour enfin permettre le déconfinement de la démocratie. Pour toutes ces raisons, c'est nous aussi aussi en toute responsabilité que nous voterons contre ce projet de loi.

Dans une situation de crise exceptionnelle, il est normal que l'exécutif dispose de moyens d'action. Ceux-ci sont considérables,

des décideurs, au sens large. Les différents groupes de notre assemblée se sont réjouis de la décision intervenue

à l'issue de débats que je qualifierai de riches et d'extrêmement condensés, des incertitudes entourent toujours la mise en oeuvre du déconfinement progressif. Mais quoi de plus normal, que nous traversons une situation aussi exceptionnelle que celle que nous vivons en ce moment ? L'exercice était inédit pour le Parlement comme pour le Gouvernement, qui devaient répondre à des questionnements fondamentaux. Comment permettre un mode de vie le plus acceptable possible dans l'attente de solutions médicales pour éradiquer ce virus qui continue à nous menacer ? Comment arbitrer entre la préservation de nos libertés et le principe de précaution ? exemple, la généralisation de l'obligation du port du masque peut être perçue comme une contrainte excessive ou comme la condition pour permettre le déconfinement. Le recours aux systèmes d'information est à notre sens utile efficace pour casser les chaînes de contamination, mais il fait dans le même temps naître des craintes légitimes quant à l'intégrité du consentement du patient et à la préservation du secret médical. La mise en quarantaine ou à l'isolement est une mesure certes protectrice, mais elle constitue dans le même temps, et de fait, une privation de liberté que nous estimons toutefois, pour notre part, correctement encadrée. Plus globalement, nous considérons que le Sénat a fourni un travail important qui a sécurisé le texte dans le respect des libertés individuelles, par exemple sur l'encadrement du délai de prorogation de l'état d'urgence sanitaire, plus respectueux du rôle du Parlement, ou encore sur la reconnaissance de la responsabilité pénale, mais aussi morale, qui pèse sur les élus à la veille de la réouverture des classes. Les garanties apportées à l'article 6 par nos commissions des lois et des affaires sociales

Cependant, nous sommes globalement convaincus que le système de traçage tel qu'il a été décidé et adopté reste un outil efficace pour contrôler la circulation du virus.

mais également la transparence des prix du matériel médical qui, nous l'espérons, va permettre à nos concitoyens d'accéder à ce matériel, notamment les masques ou les thermomètres, à des tarifs acceptables et contrôlés.

monsieur le ministre, mes chers collègues, ce que nous craignions tant a finalement pu être évité grâce aux efforts de chacun. Nos hôpitaux n'ont pas été débordés par la pandémie ; les chiffres relatifs aux contaminations et aux décès diminuent de jour en jour, et c'est heureux. Dans peu de temps, cette mesure extraordinaire qu'est le confinement sera progressivement levée. L'épidémie ralentit, mais elle n'est pas vaincue. Il nous paraît donc nécessaire de maintenir l'état d'urgence sanitaire jusqu'en juillet prochain. Dans les mois à venir, il nous appartiendra de rester sur nos gardes pour continuer à faire reculer le virus. Nos concitoyens ont majoritairement fait preuve de responsabilité et scrupuleusement appliqué les mesures barrières : ils devront poursuivre leurs efforts. l'activité du pays doit reprendre son cours. Le confinement a été salutaire, mais cette mesure ne peut durer plus longtemps sans causer des dégâts de plus en plus irréversibles, sur la santé d'abord, car bon nombre de pathologies ne sont plus traitées, sur la liberté et la justice ensuite : après avoir rappelé à plusieurs reprises que l'activité de l'administration devrait impérativement se poursuivre pour ne pas mettre en péril le fonctionnement du pays, le groupe Les Indépendants - République et Territoires se réjouit que le Sénat ait mis un terme à l'extension des délais de la détention provisoire.

Cette reprise générale de l'activité doit néanmoins être encadrée pour s'effectuer dans les meilleures conditions. Le Gouvernement dispose à présent de moyens pour mettre en oeuvre ces conditions.

L'isolement et la quarantaine sont également des outils précieux dans la lutte contre le virus. En préciser le régime était éminemment nécessaire pour limiter au maximum l'astreinte portée à nos libertés. Territoires se félicite aussi de la place faite au juge des libertés et de la détention. Le juge judiciaire est en effet l'indispensable gardien des libertés individuelles. Ses missions sont souvent accrues, il serait bon que ses moyens le soient également. La quarantaine sera également nécessaire pour enrayer la progression de l'épidémie, notamment dans les outre-mer. L'enjeu à cet égard primordial est de veiller à protéger au mieux nos territoires, dont certains ont heureusement été épargnés par le virus. C'est ainsi que sera préservée la confiance nécessaire à la reprise. Aussi centralisée que puisse être la France, la solution à cette crise ne saurait entièrement venir du Gouvernement. Beaucoup dépendra en effet de la contribution de chacun. Nous avons eu l'occasion de constater que nos concitoyens avaient su être à la hauteur de la situation. Nous leur faisons confiance pour maintenir leurs efforts. Les débats ont aussi mis en lumière le caractère incontournable des élus locaux, au premier chef desquels on trouve les maires : ce sont eux qui, sur le terrain, apportent des solutions concrètes. Il est inadmissible de leur faire courir tous les risques. Contre l'avis du Gouvernement, le Sénat a maintenu avec sagesse des dispositions visant à protéger les élus contre le risque d'un engagement de leur responsabilité pénale. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de chacun pour réussir. C'est ensemble que nous pourrons vaincre la maladie. Nous devons à nos concitoyens des mesures fortes, à la hauteur des menaces que nous devons affronter. Rien ne saurait cependant justifier le sacrifice de nos principes : dans le présent projet de loi, amendé par le Sénat, nous avons su trouver des solutions d'équilibre satisfaisantes. « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre » écrivait Dostoïevski. Nous, nous continuons à croire en des jours meilleurs pour la France et nous faisons confiance aux Français pour réussir le déconfinement. Le groupe Les Indépendants - République et

C'est tard, c'est même trop tard pour 25 000 Français ! Le peuple français est un grand peuple. Il a enduré les pires souffrances et réalisé les plus grands exploits. À travers l'histoire, il a accepté de verser son sang, sa sueur et tellement de larmes, mais à une condition que ceux qui gouvernent soient sincères, francs et courageux, que leur chef leur dise la vérité et leur montre le cap. Quand Clemenceau visitait les tranchées des poilus, il fournissait les armes, les casques et les obus pour tenir sa promesse : « On les aura Et on les a eus ! Le gouvernement actuel promet lui aussi que l'on vaincra ce virus, mais il n'est pas dans les tranchées. Il est tout au plus dans les travées des assemblées et il n'a toujours pas fourni les armes. Selon sa porte-parole, les masques étaient trop techniques pour que les Français en portent. Selon son Premier ministre, ils ne servaient à rien pour la population générale. Et maintenant, il s'apprête à infliger des amendes aux Français qui n'en portent pas. Difficile de suivre des chefs qui ne savent pas où ils vont et qui ne sont pas convaincants dans ce qu'ils font ! On a bien vu l'empressement du préfet de police de Paris de verbaliser les Franciliens qui partaient en vacances. Tout le monde s'est étonné, et même scandalisé, de ces images de banlieue sur lesquelles on voit des attaquer des policiers et des pompiers avec des cocktails Molotov, le tout dans une ambiance de capitulation médiatique et politique ! Je vous l'ai déjà dit il y a trois semaines, monsieur le ministre : vous avez menti et des Français sont morts ! Vous avez menti, et maintenant vous tremblez Vous avez peur de la réaction des Français que vous traitez comme des enfants. Vous avez peur de la justice et vous ouvrez grand votre parapluie pour vous protéger des conséquences de vos actes, en votant ici même ce nouveau concept en droit qu'est l'irresponsabilité politique. Je l'ai voté Nous sommes prêts, avez-vous affirmé, monsieur le ministre. Les Français, eux, ne le sont plus : ils ne sont plus disposés à subir les conséquences de votre impréparation et de vos mensonges. Ils ne sont plus prêts à voir l'hôpital public subir des coupes budgétaires, leurs entreprises fermer et leurs emplois détruits, leurs proches mourir et leurs anciens abandonnés par votre faute. Après nous avoir dit de rester chez nous, mais d'aller voter, vous nous dites de respecter les gestes barrières, mais de mettre nos enfants à l'école. La mort d'un adulte est une tragédie, celle d'un enfant serait un drame impardonnable ! Encore une fois, vous vous protégez en déclarant que la reprise se fera sur la base du volontariat, mais que feront

Les Français vous qualifiaient déjà d'incompétents. Il suffira d'un enfant, d'un seul enfant qui meurt du coronavirus après son retour à l'école pour que la sentence du peuple de France tombe, implacable et irrévocable : vous serez reconnus responsables et coupables d'une politique criminelle ! Je voterai bien entendu contre ce projet de loi.